L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République

La circulaire du 10 juillet 2020 prévoit d'ailleurs que, après quatre années d'expérimentation et de coconstruction, le dispositif Pix sera généralisé dans les collèges et lycées.

Je n'ai d'ailleurs personnellement aucun grief contre le principe de l'instruction en famille. Il est d'ailleurs bien possible que ce cadre puisse, dans certains cas, permettre un meilleur apprentissage. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de l'encadrer par des autorisations larges, qui permettent de préserver la liberté d'enseignement des parents l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique, mais également l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le sujet, tout autre, est celui de l'enfance et du rôle structurant de l'école au cours de cette période de la vie. L'enfance n'est-elle pas la période de la découverte des autres, de la confrontation avec des camarades différents de ses frères et soeurs sur tous les plans ?

L'enfance n'est-elle pas ce moment où l'on se confronte à une autorité, à une façon de penser différente de son père ou de sa mère ? Qui de mieux qu'un instituteur ou un professeur pour remplir ce rôle ? D'aucuns regrettent le rôle de cohésion sociale que jouait le service militaire. Mais alors, comment accepter de « zapper » l'école qui est le lieu où l'on se frotte aux autres, où l'on apprend les choses de la vie, ses règles, ses frustrations aussi ? L'école est l'apprentissage de la vie en société. Or la société n'est pas la communauté : on se socialise davantage à l'école qu'en demeurant dans le cercle familial. L'école offre l'accès à une mixité sociale improvisée, à une diversité non choisie. Creuset de la découverte, de la différence, de l'apprentissage de la vie en société, l'école permet à l'enfant de bénéficier d'une instruction partagée et ouverte sur le monde. Remettre l'école républicaine et son importance capitale au coeur des débats

vise à le rétablir dans une rédaction proche de celle qui est issue des travaux de l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste est favorable à la mise en place d'une autorisation préalable à l'instruction en famille. Ce mode de scolarisation, certes marginal,

Seule la scolarisation est garante de ces apprentissages qui, loin d'être anecdotiques, sont fondamentaux. Les contrôles de ce mode d'instruction, actuellement soumis à simple déclaration préalable, sont tout à fait aléatoires et plus ou moins mal effectués. Le dispositif prévoyant non pas l'interdiction de l'instruction en famille, comme l'avait initialement envisagé le Président de la République, mais son statut dérogatoire

Par les valeurs qu'elle véhicule, l'école est aussi le socle de notre République laïque. En deux ans, le nombre d'enfants instruits en famille a augmenté de plus de 50 %. Toutes les classes d'âge sont sont concernées. La tendance étant structurelle, il nous paraît aujourd'hui nécessaire de mieux encadrer l'instruction en famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Que nous apprennent les rapports des contrôles pédagogiques ? Que le droit à l'instruction n'est pas toujours garanti de façon suffisante ; que l'instruction en famille est de plus en plus détournée que cet éloignement peut donner lieu à des dérives sectaires, communautaires, ou alors à la mise en danger des enfants. Parmi les signalements transmis, certains relèvent des comportements très préoccupants. C'est aussi un enjeu de santé publique : dépistage des troubles, vérification du respect des obligations vaccinales, éducation à l'alimentation et à la sexualité.

L'article 21, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoyait de substituer au régime actuel un régime d'autorisation préalable de l'instruction en famille limitant son recours à quatre motifs.

de disposer d'une assise plus solide. Je ne referai l'histoire constitutionnelle ni de la liberté d'instruction en famille ni de la liberté d'enseignement. Néanmoins, comme vous le savez, lorsqu'en 1977 le juge constitutionnel a

législatifs des années 1880 montrent que l'instruction en famille n'est pas du tout partie prenante de la nouvelle logique éducative installée par les lois de la République. Au contraire, elle apparaît comme une sorte de

Nous savons qu'il y a de la bonne et de la mauvaise instruction en famille, et nous serions en tort si nous ne faisions pas la distinction entre les deux. Seront en tort tous ceux qui ne font pas cette distinction en faisant semblant de ne pas voir les problèmes. Plus de la moitié des enfants qui fréquentent les structures que nous démantelons les fréquentent sous couvert de l'instruction en famille. couvert de l'instruction en famille. Devrions-nous ne rien faire ? Que pensent ceux qui tous les jours critiquent le Gouvernement en affirmant que nous n'en faisons pas assez contre le radicalisme islamiste et qui, sur ce sujet, deviennent comme aveugles aux problèmes réels qui se posent sur le terrain ?

dans les communes, ce qui est très important dans l'élaboration des mesures de carte scolaire puisque, bien souvent- vous le savez, monsieur le ministre -une ouverture ou une fermeture de classe peuvent se jouer à un élève près.

de l'instruction en famille. Ils sauront ainsi mieux déceler les éventuels manquements ou mieux répondre aux demandes des familles, toujours dans l'objectif d'offrir à chaque enfant une instruction de la plus grande qualité possible. Quel

Enfin, nous pouvons nous interroger sur la capacité des services déconcentrés de l'éducation nationale à traiter, chaque année, quelque 50 000 à 60 000 demandes d'autorisation. Les moyens ainsi mobilisés seraient utiles pour assurer le contrôle annuel effectif de l'ensemble des enfants instruits en famille.

explication de vote. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'instruction en famille est inscrite dans le droit français depuis la loi de Jules Ferry de 1882. Elle est contrôlée et encadrée

est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il existe une relation ancienne entre la République et la nécessité d'une instruction nationale qui garantisse les droits des enfants. Dans son projet de Constitution, en 1793, Condorcet l'exprimait ainsi : « L'instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres. Ce principe a été repris dans la Constitution de 1848 que je vous cite : « L'enseignement est libre. La liberté s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et sans aucune exception. Ferdinand Buisson, auquel nous devons le mot de « laïcité », et qui est l'un des promoteurs de la loi de 1905, le disait encore plus justement en ces termes : « Dès lors que nous ne pouvons songer à reconnaître pour un futur membre de la société la liberté de se passer d'enseignement, ni pour ses parents celle de l'en priver, nous ne songerons pas davantage à une sorte de liberté d'indifférence de la part de la commune et de l'État en ce qui concerne la distribution ou la non-distribution de cet enseignement. un droit et un devoir qui sont au-dessus de toutes les libertés : c'est le droit et le devoir de l'instruction qui s'imposent au nom d'une nécessité sociale. sociale. » C'est au nom de cette nécessité sociale qu'il nous semble essentiel, aujourd'hui, que l'État puisse garantir les droits

Ma conviction intime, c'est que la coexistence de propositions éducatives variées est le signe d'une société apaisée, plurielle, moderne

vous êtes montré, depuis des mois, incapable d'étayer de manière forte la corrélation qui pourrait exister entre l'instruction en famille et la menace séparatiste. Ni l'ampleur du phénomène ni celle des dérives ou des infractions constatées n'ont été explicitées pour justifier la remise en cause d'un élément constitutif d'une liberté fondamentale, la liberté d'enseignement. C'est donc sous le coup d'une démocratie de l'émotion,

à définir cet intérêt supérieur de l'enfant. Nous passons ainsi d'un régime de déclaration avec un contrôle, que

choisir que ses enfants aillent à l'école publique ou à l'école privée, choisir pour ses enfants l'enseignement à distance ou pratiquer l'instruction en famille, toutes ces décisions témoignent d'une réflexion, d'une implication et d'un engagement. L'école est obligatoire pour tous les enfants de France, mais la liberté d'instruire son enfant en dehors des bancs de l'école, selon son choix, peut répondre à des raisons diverses, qui peuvent également aux enfants autistes qui ne peuvent intégrer l'école publique, faute de classes adaptées en nombre suffisant, ou bien parce qu'ils ont des besoins différents. Nombre d'enfants ne sont pas heureux à l'école et ont besoin de travailler à leur rythme. Certains perdent confiance en eux parce que la méthode d'apprentissage n'est pas adaptée à leurs besoins. Les enfants harcelés à l'école, qui ont la boule au ventre chaque matin, peuvent avoir besoin de l'instruction en famille, au moins pour un temps, afin de reprendre confiance en eux et de retrouver goût à la vie. L'école à la maison, ce n'est pas faire ce que l'on veut de ses enfants ; c'est faire au mieux pour ses enfants. Cela implique de connaître les attendus du socle commun, de justifier ses choix pédagogiques et organisationnels, et de montrer son attachement aux valeurs de la République. de s'investir pour le bien-être et la réussite de ses enfants. Les familles que j'ai pu rencontrer privilégiaient la culture et le sport, et leurs enfants n'étaient pas isolés. L'argumentation développée par certains de mes collègues ne tient donc pas. Ne nous trompons pas de débat ! Il ne faut pas pénaliser les 0,5 % de familles qui choisissent l'IEF, mais plutôt lutter contre les abus et le séparatisme, en renforçant l'encadrement et les mesures de suivi pour ne pas perdre l'enfant en chemin. Je crois que nous sommes tous d'accord Choisissons donc de mieux encadrer, d'accompagner, de contrôler, mais pas d'interdire ! Choisissons la confiance pour tous ceux qui en sont dignes et respectent les principes de la République

M. Daniel Salmon, pour explication de vote. Monsieur le ministre, lors de l'examen en commission, le Sénat a supprimé l'article 21 relatif à la refonte de l'instruction en famille. Cet article prévoyait de remplacer le régime actuel, soumis à simple déclaration, par une autorisation des services académiques délivrée pour une durée d'un an. Ce renversement complet de la liberté d'instruction n'a d'autre but que de faire face à une radicalisation islamique qui utilise l'instruction en famille comme un outil pour déscolariser et isoler les enfants. isoler les enfants. Lors des auditions, pour évaluer la pertinence de ce revirement, nous avons demandé à plusieurs reprises des chiffres ou un ordre de grandeur sur cette radicalisation dans l'instruction en famille. Or ni le ministre ni les spécialistes- nous sommes plusieurs à l'avoir remarqué -n'ont été capables d'évaluer réellement l'ampleur du phénomène.

pourtant lucides : l'instruction en famille peut donner lieu à un certain nombre de dérives et de pratiques sectaires antirépublicaines, qui ne sont pas uniquement le fait des salafistes. Il nous faut être vigilants et rigoureux. C'est pourquoi nous sommes favorables aux mesures qui contribuent à renforcer les contrôles de l'instruction à domicile. Nous sommes également favorables aux mesures qui visent à s'assurer que les enfants suivent un projet pédagogique sérieux et conforme à nos valeurs. Nous préférons l'encadrement plutôt que la suspicion généralisée.

explication de vote. Monsieur le ministre, je salue avec beaucoup de sincérité vote détermination, votre courage et aussi votre action

Lorsque, chahuté par quelques élèves qu'il ne parvient pas à identifier, un professeur décide de sévir contre l'ensemble de la classe, non seulement il provoque un sentiment d'injustice chez les innocents qu'il a ainsi stigmatisés et châtiés, non seulement il suscite la moquerie de ceux qui n'ont pas été démasqués, non seulement il sème la zizanie entre les vrais et les faux coupables, mais il démontre aussi, et surtout, son manque d'autorité et de crédibilité. Certes, la situation plus que préoccupante, dramatique même, de petites filles embrigadées, enchaînées spirituellement selon des préceptes totalement contraires aux valeurs de la République, mérite une réponse ferme. Au pays des Lumières, de Voltaire et de Ferry, il faut évidemment lutter contre tous les obscurantismes, mais le filet jeté à juste titre sur les islamistes radicaux grâce à cet article retient aussi à tort des milliers de familles. Avec l'article 21, vous mettez brutalement fin à des choix de vie, à un droit, à une liberté vieille de cent cinquante ans. Surtout, vous méprisez et jetez par-dessus bord une denrée sociale précieuse et devenue rare, la responsabilité parentale, car les familles qui ont décidé d'instruire elles-mêmes leurs enfants doivent assumer et assument un enseignement précis et détaillé. Les récentes- et même l'actuelle -périodes de confinement ont pu faire prendre conscience à certains parents des difficultés liées à la mission d'enseigner. Nombreux ont été ceux qui ont été soulagés de voir leurs enfants retrouver le chemin de l'école, car il est difficile d'enseigner : c'est exigeant et chronophage. Quelle injustice, donc, mais aussi quel contresens social que de démissionner- au sens propre du terme -ces parents qui ont fait le choix de la responsabilité pédagogique ! Je ne voterai évidemment pas pour le rétablissement de l'article 21.

pays avait certainement besoin de moins de garde-fous, parce que la dynamique populaire d'adhésion à l'école publique submergeait tout.

les contrôles nécessaires. Il faudra sans doute renforcer les contrôles, mais aussi réaliser davantage d'inspections. Surtout, il faut admettre qu'un certain nombre de situations relèvent davantage

pas que l'école soit nuisible à l'apprentissage de la fraternité. La fraternité, ce n'est pas préférer son frère à son cousin, son cousin à son voisin, ni son voisin à un étranger. Ce n'est même pas préférer son frère à ses camarades de classe.

système de déclaration qu'on nous propose, est un bien petit sacrifice pour défendre des valeurs comme celles de la République.

Aller à l'école, c'est d'abord être ensemble les uns à côté des autres, quelles que soient les opinions politiques, religieuses, philosophiques et les

l'instruction publique et obligatoire. Un enseignement public partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une école. » La parole est à Mme Annick Billon,

pour une grande majorité d'enfants, la possibilité d'apprendre avec des méthodes pédagogiques alternatives. Les reproches faits à l'IEF ne sont étayés par aucun chiffre ni aucune statistique. Loin de moi l'idée

situation, en plus d'être pénalisante pour l'attractivité de nos territoires, m'amène à faire ce constat, monsieur le ministre : si vous voulez éventuellement limiter le recours à l'instruction en famille, laissez ouvertes les classes et les écoles dans nos villages

organisation que personne ne peut soupçonner de mener une bataille idéologique contre les intérêts des familles -fait de cette convention, « l'enfant a le droit d'aller à l'école et le droit d'avoir des loisirs ». Le droit à une socialisation, le droit à rencontrer d'autres idées que les siennes et que celles de sa famille, le droit à se former une opinion pour devenir un citoyen, le droit à développer son esprit critique sont des droits de l'enfant.

parfois même une meilleure solution que l'école dans certaines situations qui peuvent la justifier. Nous sommes nombreux ici à être ou à avoir été maires ou adjoints en charge des affaires scolaires, et à avoir été confrontés à cette instruction en famille, à des situations très particulières- on vous l'accorde -que

à des fins tout autres, notamment pour empêcher l'éducation des jeunes filles et des petits garçons et les formater. Oui, il existe probablement de très beaux exemples- on en a tous -de familles idéales qui, alors qu'elles se sont privées de tout loisir pendant un ou deux ans, ont choisi de tout arrêter pour faire un tour du monde à vélo, en caravane, en camping-car, en bateau ou en je ne sais quoi

de loi ne porte ni sur l'école ni sur l'instruction. C'est un texte sur le séparatisme et- vous l'avez précisé dans votre propos liminaire -l'objectif du nouveau dispositif que vous proposez est de lutter contre la dérive séparatiste. C'est bien dans cette optique que nous l'avons examiné, avec beaucoup d'attention,

Oui, ce texte traite de l'école de la République : il est important qu'elle continue à rassembler le maximum d'enfants dans notre pays, même s'il y a évidemment différents moyens de le faire. Nous n'avons jamais- jamais

Je ne voudrais pas que des enfants de la République aillent à l'école coranique sous couvert d'être scolarisés à domicile ; mais c'est à vous de proposer les moyens d'éviter cette dérive sans pour autant remettre en cause une liberté fondamentale

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

En France, l'instruction en famille, à distance, aussi appelée école à la maison, est déjà encadrée par le code de l'éducation. Tous les ans, l'inspection académique vérifie le respect du droit de l'enfant à l'instruction et évalue l'acquisition progressive du socle commun de connaissances. Tous les deux ans, les familles- en tout cas celles qui ne sont pas dans les zones de non-France -sont contrôlées par la mairie, qui se penche sur les raisons les poussant à choisir ce mode d'instruction. les contrôles existent et ils peuvent empêcher les dérives islamistes ; mais la réalité, c'est que, dans 98 % des cas, la conclusion est que l'instruction en famille est satisfaisante. Monsieur le ministre, malgré vos affirmations, ce texte se trompe de cible ! D'ailleurs, à ma connaissance, aucun terroriste ni même prêcheur radical n'est le produit de l'école à la maison. 60 000 enfants bénéficient aujourd'hui de ce mode d'instruction. Parmi eux, 20 000 suivent les cours réglementés du Centre national d'enseignement à distance (CNED). Si l'on choisit l'instruction en famille, ce n'est pas pour se séparer, c'est avant tout pour sauver son enfant de la déliquescence de l'école publique, détruite par l'idéologie et le comme le handicap, la pratique d'une activité sportive ou artistique de haut niveau, l'éloignement géographique d'un établissement, mais aussi le harcèlement et la phobie scolaires. la phobie scolaires. Il convenait donc de laisser aux parents de tous ces enfants le libre choix de l'instruction en famille. Les chercheurs, professionnels de la santé, historiens et pédagogues sont tous du même avis. Il faut dépasser les amalgames et les préjugés du Gouvernement : l'instruction en famille est d'un niveau exigeant, très exigeant, mais l'éducation nationale n'admet pas que l'on vienne contester son monopole dans la production industrielle d'échec scolaire. Conforter le respect des droits fondamentaux des enfants, de la diversité et de la pleine liberté éducative, c'est aussi

des sièges sociaux des organismes privés d'enseignement à distance. Mes chers collègues, cette disposition contraignante a pour objectif d'empêcher les influences étrangères dans l'instruction des enfants et d'éviter que l'enseignement à distance ne suscite la méfiance face à de potentiels excès. C'est pourquoi je vous invite à voter cet amendement de vigilance pour une meilleure liberté d'enseignement ! Quel est l'avis de la commission de la culture

ainsi. Je trouve insensé, mes chers collègues, que vous ayez été inflexibles, irréductibles, incorruptibles, pour défendre la République dans son expression vestimentaire et textile et que l'on est au coeur du dispositif de la Nation et que des familles, volontairement, sur des critères religieux, refusent l'instruction nationale parce qu'elle est nationale, vous ne vouliez pas le voir. Je ne comprends pas votre attitude.

les mots pour conclure : « Tout Français est libre d'enseigner, mais tout Français est tenu de prouver, devant les mêmes juges et de la même manière, qu'il est capable d'enseigner ; tout Français est libre d'enseigner, mais il n'est pas libre de réclamer pour son enseignement le privilège d'être clandestin, d'échapper à tous les regards, de produire tels résultats que bon lui semble, et de se refuser à les laisser constater dans les formes que fixe la loi elle-même ; tout Français est libre d'enseigner, mais à la condition de ne pas s'être volontairement placé dans une condition qui le frappe d'incapacité légale. » La parole est

du discours des Mureaux du Président de la République, qui, lui, a bien parlé de mettre fin à l'instruction à domicile. Vous reculez, mais n'essayez pas de transformer ce recul en victoire, nous vous en empêcherons

un contrôle. Par exemple, cet amendement vise à imposer que la déclaration d'instruction à domicile à la rentrée se fasse dans un délai de huit jours. Un délai était

un délai de huit jours en cas de changement, c'est-à-dire de déménagement, de modification des modalités d'instruction, mais un flou subsistait concernant les enfants instruits en famille plusieurs années de suite.

non seulement des savoirs, mais aussi des valeurs et des principes. Elle modèle les esprits de notre plus jeune génération ; en retour, on lui doit une protection sans faille. Il est regrettable que notre école publique et nos établissements d'enseignement supérieur aient été mis de côté dans ce texte. Vous avez souhaité pointer l'enseignement à domicile sans traiter le fond du problème, les petits fantômes de la République. Certes, l'instruction à domicile est en forte augmentation, mais elle ne représente que 0,5 % des élèves français, soit 62 000 enfants. Vous me répondrez qu'aucun enfant de la République ne doit être sacrifié, monsieur le ministre. Toutefois, lorsque notre dispositif de contrôle, de suivi et d'identification présente autant de trous dans la raquette, il convient de s'atteler à les colmater, et non de déclarer forfait. Lors des débats au Sénat sur la loi pour une école de la confiance, en mai 2019, j'avais défendu de nombreux amendements visant à renforcer l'opérationnalité de l'encadrement de l'instruction

Je saisis donc cette nouvelle occasion pour vous présenter des amendements pragmatiques, fruits des nombreuses auditions que j'ai menées auprès d'élus, d'inspecteurs académiques et de familles ayant fait ce choix, pour respecter l'équilibre fragile introduit par la loi de Jules Ferry de 1882.

en famille. Ce régime intermédiaire éviterait de restreindre excessivement cette liberté, contrairement au régime d'autorisation supprimé par la commission. Cette alternative permettrait également d'inviter ces familles à formaliser leur démarche pédagogique

Quelle sera la grille d'évaluation et de validation applicable aux personnes éligibles à ce dispositif ? Les validations seront-elles automatiques au bout de deux années d'instruction en famille ? Les parents éligibles devront-ils présenter un projet pédagogique précis et complet ? Cette mesure paraît en décalage avec l'esprit général du texte. D'un côté, vous souhaitez favoriser le plus possible une instruction au sein des établissements scolaires ; de l'autre, vous voulez rendre quasiment automatique la validation des acquis pour les parents assurant cette instruction en famille.

ont déposé un dossier de recevabilité en vue d'obtenir par la VAE un diplôme ou un titre délivré par l'État. Depuis 2002, toute personne peut obtenir la totalité d'une certification grâce à la reconnaissance de son expérience, que cette dernière ait été acquise dans le cadre d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. La VAE est présente dans de très nombreux ministères : le travail, la défense, l'agriculture, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, la culture, la jeunesse, la santé et les affaires sociales, ou encore l'écologie. Dans le présent article

Par ailleurs, la VAE n'est pas automatique. Il faut déposer un dossier. Actuellement, le taux de certification des dossiers présentés, tous ministères confondus, est d'un peu plus de 60 %. La VAE ne donnera pas non plus le droit d'être enseignant, bien évidemment, car il ne s'agit pas d'un concours d'entrée dans la fonction publique. Les conditions pour enseigner, y compris dans les établissements privés hors contrat, sont encadrées par des conditions de diplômes strictes. Enfin, selon le sondage réalisé par le collectif de familles en IEF Félicia ce sont les femmes qui, à 91,7 %, assurent l'instruction en famille. La mise en place de la VAE permettrait donc de reconnaître les compétences acquises

contrôlées annuellement, que cela dépendait grandement de la relation de confiance ou de proximité qu'elles avaient instaurée avec leurs représentants locaux ou les inspecteurs académiques de leur département. Les maires ne sont pas préparés à la conduite de ces enquêtes à domicile. Aucune grille d'évaluation ne leur est fournie. Tel sera d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 207 rectifié. De nombreux élus ne s'estiment pas en mesure de pénétrer au domicile de leurs administrés pour juger

les contrôles sont un moyen pour eux de prendre la température afin de constater ou non les carences éducatives et, le cas échéant, de les déclarer. Il faut donc s'assurer que le thermomètre fonctionne correctement et que, suite au diagnostic, le traitement suive. Des inspecteurs académiques m'ont confié que le constat d'un manquement dans les acquis attendus d'un enfant ne donnait pas forcément lieu à une action pour y remédier. Des mesures doivent pourtant systématiquement être prises lorsqu'un signalement est effectué. L'objet de cet amendement est donc de clarifier un dispositif qui devrait être évident, à savoir la mise en place d'une injonction d'inscription dans un établissement public ou privé en cas de défaut évident dans les acquis attendus d'un enfant instruit en famille. Quel est l'avis de la commission de la culture

adaptée, dans un environnement propice. L'objet de cet amendement est donc de rendre systématique un dispositif déjà existant : le signalement au procureur de la République de tout refus par un parent de se soumettre à une enquête ou de tout incident lié à ce contrôle.

contrôle. En second lieu, l'article 40 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit

invité les parents d'élèves qui pratiquent l'enseignement en famille et qui ne pourraient pas continuer à instruire ainsi leur enfant à rejoindre ou à créer des établissements privés hors contrat. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une perspective accessible et réaliste.

école. Les conditions à remplir pour pouvoir ouvrir une école ont fait l'objet d'une profonde redéfinition dans la loi Gatel, qui a permis de trouver un équilibre entre liberté d'enseignement

provisoirement quitter la majorité d'idées que vous formez ponctuellement ... Au début de ce quinquennat, en 2017, il était plus facile d'ouvrir une école qu'un bar,

avec sincérité et sans flagornerie votre détermination à mieux contrôler les écoles privées hors contrat et l'instruction en famille, avec des inspecteurs formés aux différentes méthodes pédagogiques. il me semblerait utile et intéressant que la commission de la culture et de l'éducation puisse disposer chaque année d'un état des lieux du nombre de contrôles effectués, du nombre de contrôles insatisfaisants

Cette triple déclaration m'avait surpris, d'autant que le représentant de l'État responsable de l'éducation doit transmettre au président du conseil départemental la liste des enfants instruits à domicile. L'amendement de Stéphane Piednoir

Il paraît pourtant difficile de retirer ce droit avant que le représentant de l'État en matière d'éducation n'ait été informé des conclusions de l'évaluation de la situation menée par l'équipe pluridisciplinaire, telle que mentionnée à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

La procédure de l'information préoccupante est un outil essentiel dans la protection de l'enfance en danger en raison de sa facilité de mise en oeuvre. Toutefois, elle peut être détournée de sa vocation première,

peut être interprétée comme rendant automatique, dès transmission d'une information préoccupante, l'information de l'éducation nationale, ce qui peut entraîner la fin de l'instruction en famille- nous souhaitons. Il me semble que la transmission de l'information au recteur dans les seules conditions prévues à l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles est trop tardive. Cet article prévoit d'aviser le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger

et non de se limiter à une simple évaluation, à disposition des responsables de l'éducation nationale. Je préfère que l'on s'inscrive dans la logique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

Ces premiers éléments constitutifs du dossier de chaque enfant concerné pourraient également être transmis aux services académiques chargés de conduire un contrôle, ce qui permettrait à ces derniers de mieux appréhender le projet pédagogique défendu par chaque famille. De nombreux parents ont le sentiment que ces contrôles sont menés à charge et qu'ils sont trop aléatoires. Je suis intimement persuadée que l'adoption de cet amendement permettrait de rétablir un climat plus apaisé, plus constructif, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Quel

était la rapporteure. Le code de l'éducation prévoit une déclaration annuelle et par écrit pour les enfants qui poursuivent d'une année sur l'autre leur instruction en famille. Or, à chaque déclaration, il sera demandé de présenter les modalités d'organisation et

Il paraît important d'affirmer le respect des valeurs de la République au coeur de cet engagement. En effet, l'instruction doit permettre à chaque enfant de devenir un citoyen libre et éclairé

savoir « l'apprentissage de la vie en société, de l'action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ».

que les enseignements dispensés dans le cadre de l'instruction en famille soient majoritairement en français, il est également souhaitable qu'ils puissent se faire en langues étrangères ou régionales, comme cela peut être proposé dans les écoles publiques ou privées dans le cadre d'un enseignement bilingue ou plurilingue.

de la culture ? Nous connaissons tous le combat de Max Brisson pour les langues régionales et sa cohérence, pas seulement avec lui-même, mais avec d'autres aussi. Je salue son engagement. Sa préoccupation est légitime : permettre l'enseignement des langues régionales, y compris dans le cadre de l'instruction en famille, c'est aussi un enjeu de transmission du patrimoine linguistique. Notre commission y est très attachée et, de manière générale, le Parlement se mobilise régulièrement en faveur des Toutefois, il me semble que cet amendement est satisfait. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture intègre les langues comme premier domaine de compétences, notamment les langues étrangères et, le cas échéant, des Le de l'instruction en famille de novembre 2020 mentionne explicitement les langues régionales : « Objectif 2 : comprendre et s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale ».

de grilles d'évaluation, de formations ou encore de moyens. Cet amendement tend donc à prévoir le principe d'un soutien méthodologique aux maires dans l'accomplissement de l'obligation qui leur incombe de réaliser l'enquête municipale préalable à l'instruction à domicile.

En revanche, je suis d'accord avec vous, cher collègue, sur le fait que certains maires ne sont pas toujours au courant de leur rôle exact en matière de contrôle de l'instruction en famille. Cela étant, la diffusion de cette information ne relève pas du domaine de la loi : une circulaire pourrait suffire.

des cas éventuels d'enfants menacés par le séparatisme ou par toutes sortes de dérives idéologiques ou religieuses. Parce que le droit pour chaque enfant à une instruction est un droit fondamental garanti par le code de l'éducation, les pouvoirs publics ont une double responsabilité

font un premier contrôle à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction. Je propose qu'il soit plutôt effectué à partir du troisième mois suivant le début de l'année scolaire. Pour les familles qui feraient leur déclaration en fin d'année scolaire, la rédaction actuelle pourrait conduire à des contrôles en fin d'été, avant même qu'elles aient concrètement préparé

Si les parents ne remplissent pas cette obligation, ils s'exposent à des sanctions pénales. Enfin, à chaque rentrée scolaire, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation devra diffuser aux représentants de l'État dans le département le guide interministériel de 2017 concernant le suivi de l'instruction en famille. Ce guide clarifie le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l'instruction en famille. Il serait donc souhaitable qu'il puisse être diffusé dans chaque département, à chaque rentrée. L'amendement n° 247 rectifié,

M. Max Brisson. Cet amendement vise à éviter la convocation des responsables de l'enfant ou de la personne chargée de l'instruire à un entretien,

Évaluer l'instruction en dehors de l'école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l'instruction dans la famille. » Ces deux chercheuses ont accompagné des inspecteurs de l'éducation nationale lors de leurs contrôles d'un enfant instruit en famille. Voici les propos d'un inspecteur : « une des familles que j'ai visitées cette année, il y avait quatre enfants, la maman était enceinte du cinquième, elle allait accoucher peut-être un mois après que je sois allée dans la famille. Je me suis vraiment posé la question, vu que c'était elle qui faisait classe. Sur les quatre, il y en avait trois qu'elle prenait en charge, l'autre était trop jeune. Je lui ai posé la question : " Comment allez-vous faire ? " S'occuper d'un bébé plus de quatre autres à qui il faut faire la classe, c'est quelque chose de compliqué. Elle m'a dit que le père allait s'arrêter trois mois. » Même si

le recteur peut convoquer les parents de l'enfant pour « apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l'enfant à l'instruction », entre le moment où la déclaration d'instruction est déposée et le premier contrôle pédagogique.

sur la situation de l'enfant. Aussi serait-il utile que la famille sache pour quelles raisons le recteur souhaite les entendre. Par conséquent, le présent amendement tend à prévoir que la demande d'entretien du recteur devra être motivée.

Mme Véronique Guillotin. Chaque année, les parents ayant fait le choix de l'instruction en famille ont jusqu'au mois de septembre pour effectuer leur déclaration, les premiers contrôles de l'inspection académique étant effectués en général entre les mois de novembre et de février. À l'issue de ces premiers contrôles, les services de l'éducation nationale peuvent constater que des enfants ne sont ni inscrits à l'école publique ou privée ni déclarés en instruction à domicile. à domicile. Nous ne pouvons accepter que des enfants disparaissent aussi facilement de nos écrans radars. C'est notre rôle de garantir à chaque enfant une instruction digne de ce nom. Cet amendement vise donc à déclencher une enquête immédiate de l'autorité compétente pour vérifier ou guider le choix d'instruction des enfants identifiés comme n'étant ni inscrits à l'école ni déclarés en instruction en famille.

Je comprends bien la démarche de notre rapporteur, qui souhaite que tous les enfants scolarisés bénéficient d'un accès régulier à un professionnel de santé. Toutefois, tel est déjà le cas. En effet, de la naissance jusqu'à l'âge de 16 ans, vingt examens médicaux obligatoires sont prévus. Il n'est pas souhaitable que la présentation de ce certificat soit liée à l'enquête menée au sein des familles ayant fait le choix d'un enseignement à domicile. Ce contrôle vise, je le rappelle, à s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant

à un professionnel de santé. Des visites et des dépistages médicaux obligatoires dans le cadre scolaire sont également prévus à 3 ans, à 6 ans et à 12 ans. L'article 21 E vise à s'assurer que les enfants instruits en famille

je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche en maintenant un nouveau régime d'autorisation. Monsieur le rapporteur pour avis, cet amendement du groupe socialiste a donc pour objet de parachever le travail que vous avez entrepris lors de l'examen en commission, en complétant le régime déclaratif applicable à l'instruction en famille, en reprenant des dispositions prévues dans l'article 21 initial. Nous souhaitons encadrer davantage le régime déclaratif de l'instruction en famille, en prévoyant dans la loi les quatre types de situations autorisant le recours à ce mode d'instruction. Il s'agira de situations de maladie ou de handicap, des cursus artistiques ou sportifs, des éloignements dus aux situations d'itinérance de la famille et de la situation propre à un enfant. Dans ce dernier cas seulement, compte tenu du flou entourant cette situation légalement prévue, mais peu encadrée, il faut bien le dire, la famille devra présenter un projet pédagogique et justifier de sa capacité à assurer l'enseignement, majoritairement en langue française.

de dérive. De fait, pour empêcher cela, il est nécessaire que les autorités compétentes de l'État chargé de ces contrôles puissent les effectuer de manière inopinée, aux fins de remédier aux défaillances précédemment évoquées.

Tous nos enfants doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique rapproché. L'instruction est l'un des piliers de notre République et tout enfant doit avoir la chance d'en bénéficier sans entrave. Aussi, lorsqu'une famille se soustrait une seconde fois au contrôle de la Dasen, par mauvaise foi avérée ou dans une tentative de fuite,

Cet amendement vise à instaurer une présomption de bonne foi, en accordant aux personnes responsables un délai de huit jours suivant la mise en demeure pour procéder à la déclaration. Si ce

dans la famille, dans un délai de huit jours. Dans un second temps, et seulement en cas de non-respect de cette mise en demeure, il vise à mettre en demeure les personnes responsables d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. ne vont pas dans le sens du droit à l'éducation de l'enfant. En effet, le délai supplémentaire octroyé aux personnes responsables de l'enfant risque de les inciter à ne pas procéder à la déclaration d'instruction et à attendre d'être repérées et mises en demeure par les services de l'éducation nationale avant de se résoudre à l'effectuer.

Aujourd'hui, notre dispositif est loin d'être optimal, monsieur le ministre. Il serait difficile d'affirmer le contraire. Comment, dans ces conditions, faire respecter l'obligation d'instruction, comment s'assurer qu'il n'y a plus d'enfants « hors radars » ? En 2019, le Défenseur des enfants a déploré le fait que plus de 100 000 enfants

départementale des finances publiques, la caisse d'allocations familiales et la préfecture. Ces différents services assurent le suivi des enfants et ces cellules veillent à la mise en oeuvre de l'obligation d'instruction, soit dans des établissements publics ou privés, soit dans le cadre de l'instruction en famille.

de la CAF et ceux de l'éducation nationale. La mission d'information « flash » de nos collègues députées Anne Brugnera et George Paul-Langevin a montré les limites de ce dispositif,

Plutôt que d'entraver la liberté d'instruction en famille, il convient d'assurer un suivi des enfants hors système par tous les moyens possibles. De nombreux enfants sont victimes de dérives communautaristes et échappent aux radars. La déclaration du chef d'établissement permet de ne perdre aucun élève initialement scolarisé dans le cadre prévu par la loi. En effet, l'article L. 131-2 du code de l'éducation rappelle que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. Cet amendement vise à intégrer, aux côtés de l'État, le maire et les chefs d'établissement, trop souvent oubliés et démunis dans la lutte contre la déscolarisation. Il tend à garantir, sans empiéter sur les dispositions actuelles, la liberté d'enseignement, notamment l'instruction en famille. Dans le but de contrôler plus strictement les parents islamistes qui tenteraient de faire passer leurs enfants sous les radars de l'État, et au nom des droits de l'enfant, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement. Quel est l'avis de la commission de la culture

le suivi et la connaissance des enfants instruits à domicile sont clairement insuffisants. Retirés de l'école sans être déclarés comme étant instruits à domicile, absents des registres ou mal instruits, ces enfants se retrouvent parfois dans des situations à risque. C'est un fait : de trop nombreux enfants échappent encore au contrôle des services de l'État et des services sociaux. C'est pourquoi j'avais déposé, en 2019, une proposition de loi visant à renforcer l'identification, le contrôle et le suivi de l'instruction à domicile. L'article 3 de ce texte visait à améliorer le suivi et l'identification à l'échelon national des enfants non scolarisés en leur attribuant à tous un numéro d'identification national élève, le fameux « INE », dès l'âge de l'instruction obligatoire. À l'époque, cette proposition de loi, déposée également sous forme d'amendement au projet de loi pour une école de la confiance, n'avait pas suscité l'engouement que nous constatons aujourd'hui ; elle était néanmoins annonciatrice des débats que nous avons en ce moment même. Il nous aura fallu attendre deux ans

L'article 21 a été introduit lors des débats à l'Assemblée nationale ; il vient compléter le code de l'éducation d'un nouvel article prévoyant que chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction se voit doté d'un identifiant national. Cet identifiant concernera donc tous les enfants à partir de trois ans, âge du début de l'instruction obligatoire. Cet article octroie ainsi une base légale à l'actuel INE, créé par arrêté en 2012. Néanmoins, la rédaction du début de l'article nous pose problème. Un identifiant de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction ». Autrement dit, rien n'indique que cet identifiant ne sera pas utilisé

ou n'encadre ces potentielles autres utilisations de l'identifiant national. Il nous semble dangereux de laisser ouverte la possibilité d'utiliser cet identifiant pour d'autres finalités non précisées par le législateur

La suppression du terme « notamment », objet d'un débat législatif assez récurrent, limiterait l'utilisation de l'INE au seul suivi de l'obligation scolaire.

que la suppression de l'adverbe « notamment » ne permettrait plus de viser : l'INE ne pourrait plus être utilisé pour les raisons statistiques ou de gestion qui motivent son usage actuel.

je considère que c'est chose faite. Cela vaut pour ce sujet comme pour d'autres. C'est pourquoi je profite de cette intervention pour signaler l'existence de ce comité d'éthique qui fut d'abord présidé par

Delattre, pour présenter l'amendement n° 216 rectifié. La mise en place par nos collègues députés d'un identifiant national pour tous les enfants soumis à l'obligation d'instruction, y compris ceux qui sont instruits en famille, est une très louable avancée. L'INE permettra à l'évidence de mieux recenser et par conséquent de mieux contrôler les enfants qui seraient inconnus des services de l'éducation nationale, dits « hors radar

Je relève en particulier la pertinence des cellules de protection du droit à l'instruction qui, réunissant plusieurs services et pouvoirs publics, permettront un meilleur partage des informations. Dans cet esprit, nous proposons, par cet amendement, de faire inscrire au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) l'identifiant national élève prévu à l'article 21 du projet de loi. Le croisement des fichiers est un bon levier pour le repérage des enfants désengagés du système scolaire. La parole

d'égal accès à l'instruction. Les enfants déscolarisés sont difficilement identifiables et ne peuvent aisément se voir attribuer un INE. Repérer puis suivre ces enfants qui ne bénéficient pas de la moindre forme d'instruction est pourtant fondamental : la création des cellules de protection du droit à l'instruction, prévue à l'article 21 H

des enfants déscolarisés. En effet, sachant que ce dernier répertoire recense l'ensemble des enfants de plus de trois ans présents sur le territoire national au moyen de leur numéro d'inscription au répertoire (NIR), le croisement du RNIPP et des INE permettrait d'identifier automatiquement les enfants déscolarisés en repérant les enfants de plus de trois ans sans INE.

ans, a créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est précisément sur cette question du numéro universel. À chaque fois que cette idée revient dans les débats parlementaires, comptez sur des personnes comme moi pour rappeler la nécessité de ne jamais y faire

Je vous remercie

Or l'instruction est un droit qui fait partie de notre pacte républicain. Cet amendement vise donc à garantir le principe consistant à ne laisser aucun enfant sans solution scolaire. Ce dispositif prévoit pour cela, le croisement des fichiers découlant du recensement effectué par le maire et de l'identifiant national et, d'autre part, la recherche rapide d'une solution éducative. Quel est l'avis de la commission de la culture

est ainsi libellé : La parole est à Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à permettre l'entrée en vigueur, dès la rentrée 2021, de l'identifiant national attribué aux enfants instruits en famille. Pour rappel, le numéro INE a été mis en place il y a plus de quinze ans, 26 millions d'identifiants ont déjà été créés et son système d'information est d'ores et déjà opérationnel. Le chantier INE pour tous est donc largement entamé. Nous corrigeons ici les angles morts qui demeurent, soit les enfants des premier et second degrés de l'enseignement privé hors contrat, ainsi que les enfants instruits à domicile. Il s'agit donc d'une minorité d'élèves : on parle de 125 000 nouveaux numéros à créer.

Christian Bilhac. L'article L. 111-1 du code de l'éducation rappelle, dans une rédaction dense, le rôle fondamental de l'éducation et le droit intangible à l'instruction pour tous les enfants. Le deuxième alinéa de cet article dispose : « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Cet amendement vise à préciser davantage cette phrase. Tout d'abord, il s'agit de reprendre l'intitulé exact du décret du 31 mars 2015 qui mentionne « un socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». Nous préférons cette dernière phrase à l'expression « transmission des connaissances », qui est limitative. Ensuite, toujours au sein de cet article L. 111-1, nous voulons décliner précisément les valeurs de la République pour rappeler expressément que nos enfants devront s'approprier dès l'école les notions de liberté, d'égalité et de fraternité. J'ajouterai que ce socle ainsi clarifié devra, par ailleurs, être partagé par l'ensemble de la communauté éducative au sein de l'école publique

des valeurs de la République ne suffit-il pas ? La présidente du Conseil supérieur des programmes nous a dit la semaine dernière que la transmission des connaissances ancrées dans les disciplines au coeur des programmes

à Mme Nathalie Delattre. Comme je l'ai souligné lors de la présentation de l'amendement n° 213 rectifié, lorsque les maires effectuent des contrôles au sein du domicile des familles ayant fait le choix de l'instruction en famille, ils ne disposent pas des outils nécessaires pour les mener dans de bonnes conditions. Comment pouvez-vous demander à un élu local de mener des contrôles sans que celui-ci puisse se baser sur des critères définis, objectifs et partagés par tous, et sans qu'une grille d'évaluation lui soit fournie pour une enquête utile et documentée ? Les maires se sentent désemparés face à cette situation. Bon nombre d'entre eux ne sont pas à l'aise à l'idée d'effectuer ces contrôles. Ils ne s'estiment pas les plus à même pour le faire. À cela s'ajoute le sentiment d'intrusion que peuvent provoquer ces enquêtes au coeur du domicile familial. Il est impératif de leur donner les moyens de les mener dans les meilleures conditions. Nous nous devons de les accompagner. Dès lors, nous pourrions mettre en place une grille d'évaluation pour les maires lorsqu'ils doivent conduire cette enquête sur l'instruction en famille. Il s'agit de leur donner un cadre et d'établir des critères d'évaluation précis. Cela leur permettrait, à l'issue de l'enquête, de déterminer si les enfants suivent ou non l'enseignement à domicile dans un environnement propice et dans de bonnes conditions.

Le code de l'éducation prévoit déjà un dispositif de contrôle pour vérifier la situation scolaire des enfants. Ces contrôles associent les collectivités locales et les services de l'éducation nationale, et peuvent aller jusqu'à des mises en demeure de scolariser un enfant. Tous ces pouvoirs publics font du mieux qu'ils peuvent, mais nous devons aller plus loin aujourd'hui compte tenu de la forte progression des déclarations d'instruction en famille et de l'émergence, depuis quelques années, des écoles « de fait ». À bien des égards, le projet de loi enrichit les possibilités d'identifier les enfants que l'on suppose hors radars et potentiellement sous emprise idéologique. Je pense, en particulier, à la mise en place de cellules de protection du droit à l'instruction, qui est une bonne mesure. En parallèle, cet amendement déposé par Christian Bilhac vise à responsabiliser les familles en conditionnant le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la présentation d'un certificat de scolarité. Outre la pression que pourrait exercer cette mesure sur les familles, il est souhaitable de s'assurer qu'une aide sociale est bien utilisée conformément à

Le code de la sécurité sociale conditionne en effet le versement de cette allocation, et plus largement des prestations familiales, à la présentation des justificatifs d'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire ou d'instruction dans la famille pour certaines prestations. La loi fait donc obligation de s'assurer que les exigences prévues en termes d'instruction des enfants sont respectées pour verser aux familles l'allocation de rentrée scolaire et les autres prestations familiales. Il leur appartient également de suspendre le versement des prestations en cas de non-présentation de ces documents jusqu'à ce qu'ils soient transmis.

et que l'on est en âge de voter. Or ce n'est vrai qu'en partie. La citoyenneté, ce sont des valeurs, des droits et des devoirs qui se transmettent dès le plus jeune âge. En ce sens, les conseils municipaux des enfants sont un excellent moyen de faire découvrir nos institutions et nos principes républicains tels que la laïcité. Le parlement des enfants regroupe 577 classes de CM2, toutes invitées à participer à une leçon d'éducation civique grandeur nature. Nous comptons également près de 1 300 conseils d'enfants animés par 25 000 enfants âgés de 7 ans à 8 ans. J'ai pu constater dans mon département l'enthousiasme de ces enfants, qui font partie de laboratoires d'idées censés représenter l'ensemble des jeunes de leur classe d'âge et du territoire concerné. Il est difficile cependant à ces structures d'être véritablement représentatives lorsque vous en excluez les enfants en instruction en famille. Nous ne pouvons pas

comme leurs camarades en école, à l'exercice de leur citoyenneté au sein des conseils municipaux ou des parlements des enfants. Quel

l'amendement n° 107 rectifié. Cet amendement a pour objet de soumettre l'ouverture des établissements d'enseignement privés hors contrat, actuellement soumis à simple déclaration, à un régime d'autorisation d'ailleurs en vigueur en Alsace-Moselle depuis 1873. Je rappelle que ce souhait d'établir un régime d'autorisation préalable répond à une préoccupation ancienne et constante de notre groupe. Nous avions essayé de l'instaurer en

leur création. Il existe environ 1 600 établissements scolaires hors contrat sur les 9 700 écoles privées. Leur nombre croît chaque année, ce qui est extrêmement inquiétant, quand on sait que les services de l'État reçoivent des signalements de plus en plus nombreux pour insuffisance ou absence d'instruction, ou pour non-adéquation de celle-ci avec les principes de la République, mais aussi pour utilisation de locaux non adaptés à l'enseignement, voire insalubres. Surtout, de très nombreux phénomènes de radicalisation et de sectarisme, ainsi que des problèmes pédagogiques, sont dénoncés au sein de ces écoles. Le régime d'autorisation que nous proposons permettrait un contrôle renforcé aussi bien administratif et financier que pédagogique. Il permettrait également un véritable dialogue en amont entre l'administration et les porteurs de projets, ce qui éviterait d'éventuels problèmes et des situations dangereuses ou des contentieux ultérieurs de nature à nuire à l'intérêt ou à la santé des enfants scolarisés dans ces établissements. Ce dispositif constituerait, en outre, le corollaire du régime d'autorisation pour dispenser l'instruction en famille, qui pourrait être bientôt requis si l'article 21 du projet de loi était rétabli- sait-on jamais -au cours de la navette parlementaire. La parole est à M. Pierre

Je vous rappelle encore une fois le texte de la Constitution du 4 novembre 1848 : « La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois. » C'est tout à fait fondamental

Avec Tocqueville, vous vous rattachez à une démocratie libérale, qui considère que la famille a des droits sur l'enfant supérieurs à ceux de la Nation. Avec la République, nous défendons le contraire. Nous considérons que la Nation, parce qu'elle a un objectif d'instruction nationale,

outre, les modalités de contrôle des écoles hors contrat ont été renforcées. Ainsi, tous les établissements hors contrat font l'objet d'un contrôle lors de leur première année d'existence. Le projet de loi que nous examinons vise également à renforcer les obligations pesant sur les établissements hors contrat. Pour toutes ces raisons, il est proposé

Il acceptera que nous fassions preuve de la même constance et que nous nous cramponnions à l'excellente loi Gatel. Quant à Pierre Ouzoulias, je l'ai connu plus inspiré.

non pas créer une autorisation d'ouverture, mais laisser les établissements s'ouvrir et ensuite les contrôler. Vous ne pouvez donc pas nous dire aujourd'hui que, grâce à cette loi, vous avez empêché l'ouverture d'établissements scolaires privés hors contrat

je ne pense pas que souhaiter une éducation émancipatrice revienne à favoriser un quelconque régime totalitaire ! Mon cher collègue, vous avez parlé de Dieu. La référence de Tocqueville est bien celle-là, en effet !

Mme Céline Brulin. Les écoles privées sous contrat sont soumises au respect des programmes de l'éducation nationale et font l'objet d'inspections régulières par l'inspection académique.

que cette formation devrait être dispensée par l'éducation nationale, puisqu'elle s'adresse à des agents qui ont pour mission d'enseigner les programmes de l'éducation nationale. De la même manière, nous pensons que l'argent public ne doit pas servir à financer tout ou partie d'une formation délivrée par un organisme confessionnel, ou dont le contenu serait

l'intitulé d'une formation au module spécifique sur le projet éducatif de l'enseignement catholique, dispensée par l'Institut normand de sciences religieuses (INSR). Cette aux professeurs stagiaires du primaire et du secondaire, toutes disciplines confondues, qui ont réussi leur concours et sont en année de titularisation. L'objectif général de cette formation donner des bases culturelles et théologiques permettant de mieux comprendre la foi chrétienne et d'éclairer le projet éducatif de l'enseignement catholique. Je vous ferai grâce de l'ensemble du contenu de ce module, mais voici tout de même un petit florilège : « Introduction à la lecture de la Bible

Pour rappel, ces établissements sont certes associés au service public de l'éducation nationale, mais ils ont le droit de conserver leur caractère propre, principe qui n'a jamais été remis en cause au cours de quelque audition que ce soit. Ce droit leur a été expressément reconnu par le Conseil constitutionnel.

sein de cet enseignement catholique sous contrat, exercent des professeurs ou des apprentis professeurs qui ne sont pas catholiques et qui sont même athées. Ils ont parfaitement le droit d'enseigner dans ce type d'établissements, car il n'y a pas de discriminations

décidée par l'autorité administrative, et donc en l'absence de décision de justice, soit uniquement temporaire. Certes, il est essentiel de permettre la fermeture rapide d'un établissement privé du premier ou du second degré ou de l'enseignement technique qui ne répondrait pas à l'obligation de déclaration. Toutefois, il est également essentiel que la restriction d'une liberté fondamentale, la liberté d'enseignement, fasse l'objet d'un examen par la justice, et non uniquement par les préfets des départements après avis de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. L'amendement n° 5 rectifié, présenté

en place par la loi Gatel. À mon sens, ces alinéas ne sont pas une entrave à la liberté d'enseignement, mais un moyen de lutter contre la fraude manifeste et le non-respect volontaire des lois de la République. là du cas d'une école qui aurait ouvert quelques jours trop tôt avant le terme du délai de trois mois entre la déclaration et la possibilité d'ouvrir. Il s'agit du cas d'une ouverture sans aucune démarche, et donc sans aucune possibilité de vérification par le maire, le préfet ou le recteur de l'identité et de la compétence du chef d'établissement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou du fait que le projet éducatif correspond bien à ce que l'on peut attendre d'un établissement scolaire.

relatives aux établissements recevant du public- quelquefois pour des raisons d'hygiène -ou, dans le contexte actuel, pour non-respect des consignes sanitaires. Je demande donc le retrait

le directeur de l'établissement pourra saisir le juge administratif d'un référé liberté, procédure très rapide et réactive. Certes, la liberté d'enseignement est une liberté fondamentale, mais le droit de l'enfant à l'instruction est également garanti par la Constitution. s'agit donc d'un équilibre entre deux droits et libertés protégés par la Constitution. La fermeture administrative est possible pour ce qui concerne l'exercice d'autres libertés fondamentales, comme la liberté d'entreprendre, avec la fermeture administrative d'un établissement commercial par exemple.

en matière de libertés. Ce serait faire injure au juge administratif que de dire qu'il ne protège pas les libertés, alors qu'il porte une extrême attention à nos actions dans ce domaine comme en d'autres. La protection des libertés existe bel et bien, mais pas au détriment de l'efficacité,

les enfants ... Qu'il faille lutter contre des écoles souterraines, clandestines, je n'en disconviens pas. Mais ne les appelez pas établissements privés hors contrat ! Je maintiens donc mes amendements, même si je dois être seul à les voter.

des enfants sont les victimes de personnes malveillantes et mal intentionnées, qui créent une école privée hors contrat à de mauvaises fins.